J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires et de la proposition de loi organique relative à la nomination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

nous semble en effet tout aussi indispensable de protéger et d'investir dans les lignes capillaires, qui sont essentielles pour un aménagement harmonieux et équilibré du territoire. Elles permettent de développer les circuits courts et de renforcer la compétitivité des entreprises sur les territoires.

95 % sont imputables à la route. Faut-il continuer en ce sens ? C'est donc bien l'ensemble de nos territoires qui ont besoin d'une meilleure desserte pour le transport de marchandises par voie ferrée ou fluviale. À ce titre, les sommes prévues nous semblent largement insuffisantes. Un milliard d'euros en cinq ans, c'est seulement 200 millions d'euros par an. Lorsque l'on connaît les enjeux et surtout le potentiel de développement de ces modes de transport, c'est absolument déraisonnable. Des efforts importants doivent être faits par les pouvoirs publics pour organiser la présence non pas sur les seuls axes stratégiques, mais bien sur l'ensemble du territoire de dessertes ferrée et fluviale pour le transport de marchandises, afin de respecter les engagements pris lors de l'accord de Paris et d'engager la lutte contre les fractures territoriales.

Le développement du transport ferroviaire est évidemment un objectif très important, notamment pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Il passe par plusieurs types d'investissements. Le premier vise à remettre notre réseau ferré en état. Cela ne figure pas dans la programmation des infrastructures, puisqu'il s'agit d'investissements de SNCF Réseau. Mais, je le rappelle, grâce au nouveau pacte ferroviaire, nous avons décidé d'investir 3,6 milliards d'euros par an

qui doivent faire l'objet d'investissements spécifiques. Ce n'est évidemment pas du tout contradictoire avec la remise en état de notre réseau ferré ou la politique que nous menons par ailleurs

: La parole est à M. Bruno Gilles. La réalisation de la ligne ferroviaire transalpine Lyon-Turin, qui verrait le jour à horizon 2030, serait bien entendu un atout incontestable pour le développement des échanges entre l'Italie et les pays situés à l'est de Turin et le nord de la France. Mais le sud de la France et les pays de l'arc méditerranéen pourraient être très pénalisés. Ce tunnel transfrontalier nécessitera des voies d'accès françaises, mais aussi des voies pour fluidifier le noeud ferroviaire lyonnais et desservir les deux portes d'entrée maritimes françaises, au nord et au sud, et ainsi permettre un accès fluide à l'. À ce jour, seul le barreau nord du contournement de Lyon dispose d'un tracé définitif et d'une déclaration d'utilité publique. La réalisation du barreau sud est, dès lors, très incertaine. Nous ne pouvons pas l'admettre tant cela mettrait en péril l'activité de la place portuaire de Marseille-Fos, qui se verrait notamment privée des flux en provenance d'Asie. L'absence ou le retardement du barreau sud-est aurait des conséquences désastreuses pour l'ensemble des territoires situés au sud de Lyon, qui ne seraient plus directement desservis à terme. Cette perte de trafic pour le port de Marseille-Fos s'effectuerait au profit des ports italiens, notamment Trieste. À l'heure où la Chine s'apprête à signer des accords importants avec l'Italie dans le cadre des nouvelles routes de la soie, il faut veiller à ne pas aggraver les difficultés à venir. Afin que cet axe Lyon-Turin ne fragilise pas la compétitivité des régions du sud et qu'un équilibre entre le nord et le sud de la France subsiste, il est indispensable que le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise soit total et que les barreaux nord et sud soient réalisés concomitamment. concomitamment. Le texte dont nous débattons ces jours-ci doit intégrer de tels engagements. C'est l'objet de l'amendement n° 206 rectifié, que nous sommes très nombreux à défendre sur ces travées.

qu'il porte une ambition forte en la matière et qu'il veut conforter nos places portuaires dans la concurrence mondiale. Mais, encore une fois, aucune mention n'est faite du transport de fret par wagon isolé. Pourtant, quasiment abandonné par la SNCF, le wagon isolé jouait et peut encore jouer un rôle fondamental dans l'animation du réseau fret sur l'ensemble du territoire. C'est pour cela que, depuis de nombreuses années, les sénateurs du groupe CRCE ont lutté contre un tel abandon, puis pour la relance de l'activité. Il s'agit non pas d'une lubie ou d'un entêtement dogmatique, mais bien d'un impératif économique et environnemental. Ainsi, en France, selon des chiffres du service de l'observation et des statistiques du ministère de l'environnement, l'activité wagon isolé totalisait en 2015 entre 200 000 et 250 000 mouvements de wagons chargés ou vides après avoir atteint un million de mouvements dans les années quatre-vingt-dix. À ce jour, plus de 300 gares de fret et sept grands sites de triage à la gravité ont été fermés. Ce désengagement de la SNCF a entraîné une grave dégradation du maillage ferroviaire, déjà largement amorcée, et a laissé des territoires entiers et de nombreuses PME sans solution. Pourtant, les autoroutes ferroviaires n'ont de sens que si l'on relance parallèlement le wagon isolé. Certes, le wagon isolé représente un effort logistique supérieur à un train entier ; il nécessite plus de personnels et de moyens. Mais, d'un point de vue écologique et d'aménagement du territoire, il s'agit d'un outil indispensable pour freiner l'essor constant des camions sur le réseau routier. Cela dépasse la rationalité économique. C'est pourquoi la relance du fret passe aussi, à notre sens, par la relance du wagon isolé, qui est à même de répondre aux exigences et à l'explosion du commerce en ligne. Cela suppose un investissement massif dans l'appareil de production- je pense aux infrastructures, aux chantiers de fret,

gérer au mieux leur activité et trouver les bonnes solutions opérationnelles. L'objectif est clair : redresser le fret ferroviaire et lui redonner la place qu'il doit avoir au moment où nous souhaitons tous lutter contre le changement climatique. Le Gouvernement

dans le cadre de la programmation des crédits figurant dans le rapport annexé et des contrats de plan qui les déclinent, de permettre aux collectivités locales de connaître les calendriers prévisionnels de réalisation de chaque ouvrage retenu.

Ces calendriers figurent dans l'exposé des motifs. Le Conseil d'orientation des infrastructures, le COI, précisait lui-même qu'il convenait de garder de la souplesse pour des investissements par nature potentiellement mouvants et soumis à un grand nombre d'aléas. Il paraît évident que toutes ces opérations doivent être menées en concertation avec les collectivités concernées. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement Gouvernement ? Cet amendement me paraît satisfait, puisque l'exposé des motifs précise bien les principales phases des opérations retenues dans le cadre de la programmation.

d'interconnecter les grandes métropoles du Sud-Ouest européen, mais aussi, et surtout de renforcer les modalités du quotidien pour les territoires périurbains comme pour le réseau des villes moyennes, qui, par le développement des TER, verront une offre de mobilité accrue.

du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, qui est en train de s'achever, pour un coût de 1,8 milliard d'euros. Au-delà de la région Occitanie, cette ligne répond aux enjeux de développement et d'aménagement de la France et de l'Europe, en permettant une interconnexion des lignes à grande vitesse françaises et espagnoles.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

Le Parlement européen a voté à l'unanimité le 22 novembre dernier l'intégration de la section Bordeaux-Toulouse au corridor Atlantique du réseau prioritaire européen de transport. Cela rend Cela rend cette section éligible au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le MIE 2, qui est doté de près de 30 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Il en est de même pour la section Toulouse-Narbonne, qui doit être rattachée au corridor méditerranéen. Ces décisions de principe doivent maintenant être concrétisées par une base légale, légale, au travers de la définition d'une structure de portage, qui pourrait prendre la forme d'une société de projet, comme cela est précisé dans l'exposé des motifs du projet de loi. J'insiste, car nous ne pouvons plus attendre

Elles commencent donc à réfléchir, mais elles ont besoin d'un outil, à savoir d'une société de projet. En accordant cette possibilité, vous apportez les garanties et le soutien nécessaires à l'Europe et aux collectivités territoriales. J'ajoute que cet amendement est cohérent

de développement du territoire. Ces deux projets de ligne à grande vitesse, ou LGV, en Occitanie doivent s'inscrire dans des calendriers réalistes et dynamiques. À cette fin, la reconnaissance par l'État de l'importance de ces nouvelles lignes ferroviaires permettra de concrétiser ces projets

Après dix ans d'études et de procédures, après la réaffirmation de son caractère européen, après les nombreux engagements de l'État, après l'avis du Conseil d'État du 11 avril 2018,

afin de maximiser les possibilités de cofinancement européen au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Cet amendement vise à rappeler ce principe, au regard des conditions d'application du mécanisme précité.

pourrait permettre le quasi-doublement du trafic ferroviaire des voyageurs entre la France et l'Espagne, qui passera de 4,6 à 8,8 millions de voyageurs par an.

ne présente pas en effet des avantages comparables aux lignes projetées ». Conformément aux conditions d'application du mécanisme d'interconnexion pour l'Europe, une part de financement de 20 % est attendue de l'Union européenne pour les deux branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Ce taux de financement pourrait être porté, au moins en partie, à 40 % pour la section Dax-Espagne si son caractère européen et transfrontalier était avéré.

Ces demandes de calendrier sont satisfaites par la référence au tableau du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, le COI, que nous avons introduite sur l'initiative de notre collègue Rémy Pointereau en commission

Enfin, s'agissant de la ligne Bordeaux-Dax, des travaux d'amélioration à hauteur de 500 millions d'euros sont prévus, avec pour objectif prioritaire de développer le fret ferroviaire. Tous ceux qui habitent

Le prochain cadre financier pluriannuel couvrira la période 2021-2027. » Par ailleurs, en décembre, le Parlement européen a adopté son rapport proposant d'ajouter le chaînon manquant Montpellier-Perpignan, mais aussi les liaisons Bordeaux-Toulouse et Toulouse-Narbonne. Cette inscription dans les lignes prioritaires suffira-t-elle à relancer le projet ferroviaire en Occitanie ? Comme le faisait remarquer un journaliste,

brique indispensable pour que des financements européens puissent être débloqués. Ne laissons pas passer cette possibilité, faute de quoi tout serait remis aux calendes grecques, ce qui serait désastreux ! Je le répète, l'enjeu est local, régional, national, européen. Nous parlons là de véritables leviers économiques pour l'eurorégion, qu'il s'agisse du chaînon manquant Montpellier-Perpignan ou des liaisons Bordeaux-Toulouse et Toulouse-Narbonne. J'insiste, il importe d'ouvrir les portes de la plus grande région de France sur l'Europe et sur l'Espagne.

Notre devise, madame la ministre, en ce domaine et sur ces deux dossiers, est : « un pour tous et tous pour un

à finaliser le projet Paris-Montpellier-Barcelone-Madrid. N'oublions pas que ce tronçon a été jugé comme hautement prioritaire en 1994.

clairement mentionnés dans l'exposé des motifs. Ils font même partie des rares projets pour lesquels il est proposé de continuer de travailler avec les collectivités concernées, afin d'accélérer le calendrier

L'ensemble de ces projets est intégré dans la programmation selon le calendrier proposé dans le scénario 2 du Conseil d'orientation des infrastructures. Voilà pourquoi j'ai demandé le retrait de ces amendements. C'est le Parlement

iront tout d'abord aux grands projets ferroviaires, et notamment aux lignes nouvelles. » Le premier projet cité est le Grand projet du Sud-Ouest : « Les travaux seront lancés dans la période 2018-2022.

Dans l'esprit des accords internationaux, la réalisation de ces accès était la contrepartie d'une contribution financière plus élevée de l'Italie au tunnel de base. S'agissant des voies d'accès au tunnel, le rapport du COI a proposé de repousser les aménagements aux calendes grecques.

Ces 700 millions d'euros seraient donc bien mieux utilisés s'ils étaient consacrés au projet initial des voies d'accès. Surtout, et j'y insiste, cet amendement a pour objet de rassurer nos partenaires italiens et de l'Union européenne dans un contexte très délicat.

Enfin, ce projet international présente un intérêt territorial en contribuant à la mobilité du quotidien des citoyens l'amélioration des dessertes ferroviaires entre Lyon et les métropoles du Sud alpin, Grenoble, Chambéry et Annecy.

entre Lyon et la section transfrontalière du tunnel. Ce rapport devra comprendre le phasage des travaux et leur financement précisément définis, dans la perspective de la mise en service de ce tunnel prévue en 2030. » Cela va beaucoup plus loin que ce que prévoit

que présente ce projet pour l'aménagement du territoire », en considérant notamment que « l'aménagement des lignes ferroviaires existantes entre Bordeaux et Dax [ ...] ne présente pas en effet des avantages comparables aux lignes projetées. » Cette option de programmation tend dès lors à construction d'une grande voie de communication européenne, alors même que celle-ci fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique publiée au le 5 juin 2016 pour quinze ans, soit bien avant l'échéance de de 2037 prévue dans le cadre de la programmation d'investissement. C'est pourquoi le calendrier de programmation doit pouvoir faire l'objet d'une actualisation, afin qu'il ne soit pas fait d'impasse landaise

chose, monsieur le rapporteur.

Les habitants n'en peuvent plus ! Pourtant, tout est prêt. Le tracé est adopté depuis 2009, l'utilité publique est acquise depuis 2012 et la clé de répartition des financements entre les financeurs est définie.

Alors que la première phase de ce projet a abouti avec succès en 2011, la seconde a été, quant à elle, maintes fois reportée. On parle maintenant d'un achèvement en 2038. Ce projet présente pourtant un double enjeu de mobilité. D'abord, un enjeu de mobilité nationale : il s'agit de la première ligne à grande vitesse de province à province et d'un projet contribuant à la décarbonisation des transports sur un axe caractérisé par des déplacements massifs par la route. européen : ce projet s'inscrit dans le plan de travail du corridor mer du Nord-Méditerranée et s'avère essentiel pour l'interconnexion ferroviaire en Europe. D'intérêt général, cette ligne à grande vitesse, une fois achevée, couvrira pas moins de 10 % du trafic TGV national et desservira 32 destinations, dont 8 à l'étranger. À l'heure actuelle, les usagers dénoncent une desserte incomplète et surtout incohérente. Économiquement, le projet est rentable et utile pour la collectivité, mais sa pleine rentabilité ne sera atteinte qu'avec la réalisation de la seconde phase. Financièrement, des pistes d'optimisation ont été identifiées en 2016, permettant de réduire le coût global des travaux de la section de plus de 160 millions d'euros pour un coût désormais établi à moins de 700 millions d'euros. La part de l'État ne représenterait que 200 millions d'euros, les collectivités se disant prêtes à assumer une part beaucoup plus importante. Madame la ministre, après la suppression des trains de nuit, le report aux calendes grecques d'un projet essentiel à la desserte nationale comme européenne ainsi qu'à l'attractivité de nos territoires serait une grave erreur. C'est pourquoi je vous propose d'inclure l'achèvement de cette ligne dans le projet de loi et de poursuivre le dialogue avec les collectivités concernées pour avancer. La parole est à M.

à la veille des élections européennes. Alors que le Président de la République, qui vous a nommée dans votre ministère, vient de parler de l'importance de l'Europe, le développement de cette ligne européenne est fondamental. Les lignes européennes ne passent pas toutes par Paris. L'axe Francfort-Barcelone transite par la vallée du Rhin et celle du Rhône. C'est dans ce sens que les collectivités locales se sont engagées, par un protocole que j'ai signé en tant que président de la communauté urbaine en 2012, à payer 50 % de la seconde phase.

alors que 82 millions d'euros ont déjà été dépensés pour les études de la seconde phase, est une aberration économique, une aberration européenne et une aberration au regard des engagements pris dans le cadre du plan Climat. Si nous voulons, au sein de l'Europe,

cela est rappelé dans le rapport, ne vise aucun projet qui ne soit pas hexagonal. Or nous devons penser européen, et c'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers collègues, de soutenir cet amendement.

d'évaluer les différents projets et calendriers de travaux. La loi ne saurait figer ces éléments pour des raisons que j'évoque depuis hier. Je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements,

Cela montre les limites d'un exercice qui consisterait à faire figurer certains projets dans le rapport annexé plutôt que dans la liste que votre commission a décidé d'annexer au projet de loi.

Cela étant dit, l'étude qui a été menée par le COI conclut à la nécessité d'optimiser l'offre sur la ligne existante avant d'envisager la réalisation du prolongement de la branche est de la LGV

C'est le cas de la branche est du TGV Rhin-Rhône. Faites bien attention à cette parole de l'État qui est en permanence remise en cause ... Comme vient de le dire mon collègue Martial Bourquin, la seconde

possible des moyens nécessaires et suffisants- c'est ce que nous avons tenté de faire dans ce texte -pour financer l'ensemble de ces projets. Il faudrait 1 milliard d'euros supplémentaire chaque année pour y parvenir.

il appartiendra au Gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances, de donner éventuellement une orientation en ce sens, de trouver les ressources pour permettre à l'ensemble de ces projets d'être réalisés dans les meilleurs délais. Ma position en tant n'est pas forcément très confortable, parce que je dois donner des avis défavorables à tous ces projets pour être cohérent avec, à la fois, la position de la commission et les orientations stratégiques que nous avons définies. Vous êtes évidemment libres, mes chers encore approuver d'autres projets. Nous en avons rejeté un certain nombre hier et aujourd'hui- dommage pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier d'un vote favorable. Mais cet inventaire à la Prévert

vote. Je voterai ces amendements, car je considère qu'en l'état actuel du texte la masse des investissements prévus pour l'ensemble du secteur ferroviaire n'est pas suffisante.

Vous savez donc que les travaux de la mise à 2x2 voies de la route nationale 141 ne sont pas terminés, même s'ils avancent, et qu'une dernière section doit encore être programmée dans un futur contrat de plan État-région.

est financé à hauteur de 112 millions d'euros pour la section Exideuil-Chasseneuil, entre Limoges et Angoulême, et de 40 millions d'euros pour la section La Vigerie-Villesèche, entre Angoulême et Cognac. Le contrat de plan prévoit donc une enveloppe de 150 millions d'euros

J'ai demandé au préfet de Nouvelle-Aquitaine de réunir de nouveau tous les acteurs concernés pour définir une stratégie d'action, afin d'assurer la pérennité de cette ligne. Madame

Tout simplement parce qu'il reste 70 kilomètres de route nationale qui traversent de nombreux villages, avec les risques que cela comporte. Les riverains subissent un défilé incessant de véhicules sous leurs fenêtres : 16 000 voitures- 25 000 lors des départs en vacances -et 1 000 poids lourds tous les jours. Qu'a-t-on fait ces dernières années ? Un traité international, signé en mars 2017 par Bernard Cazeneuve, prévoit d'améliorer la viabilité hivernale de cet axe de circulation avec la création de paravalanches entre Ax-les-Thermes et la frontière andorrane et un investissement conjoint des deux pays, ce qui est une première en matière d'axe routier. L'État, quant à lui, est aussi partie prenante dans une convention conclue avec le conseil départemental de l'Ariège et le conseil régional d'Occitanie qui se sont engagés à cofinancer les travaux, afin d'améliorer les conditions de circulation sur cette partie de la route nationale 20 par la création de contournements de certaines villes, notamment de Tarascon-sur-Ariège, et par l'aménagement de nouvelles voies de dépassement. Il ne s'agit pas, comme vous pouvez le constater, madame la ministre, d'un projet de 2x2 voies. Près de deux ans jour pour jour après la signature de ces deux textes, où en est-on ? Alors que tout est prêt, même terminé côté espagnol, nous produisons des études, voire des études d'études, mais toujours pas de chantier engagé. Les Andorrans ont inscrit 10,5 millions d'euros dans leur programmation budgétaire de 2018 et ne comprennent pas ces lenteurs. La région Occitanie et le département de l'Ariège ont clairement affiché leur engagement financier à hauteur de 135 millions d'euros. Nous attendons maintenant celui de l'État, afin de matérialiser rapidement les engagements pris en mars 2017 pour accélérer le calendrier de la modernisation et de la sécurisation de cette cinquantaine de kilomètres de l'axe Toulouse-Barcelone. Quel est l'avis de la commission

hier soir, même s'il est toujours important de dire combien nous sommes attachés au fait que la seule route nationale qui traverse notre département de l'Ardèche, et qui

entre les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, maillon essentiel de l'axe routier majeur entre le nord et le sud de l'Europe. En effet, il ne figure pas dans la programmation du scénario 2 proposé par le Conseil d'orientation des infrastructures, qui fait référence dans le rapport annexé au présent projet de loi. Depuis 1987, date de l'annonce d'une autoroute entre Grenoble et Sisteron, les décisions gouvernementales n'ont pas permis de finaliser cette liaison, pourtant stratégique, visant à délester la vallée du Rhône, à relier les Alpes du Nord aux Alpes du Sud et à réaliser une continuité autoroutière entre la mer du Nord et la Méditerranée. L'inclusion de l'achèvement de l'A 51 entre le col du Fau, dans l'Isère, où elle arrive actuellement, et les Hautes-Alpes, est parfaitement cohérente avec les objectifs du projet de loi d'orientation des mobilités. En effet, cet aménagement, d'une longueur inférieure à 100 kilomètres, contribuera à finaliser un grand itinéraire routier. Il participera à fluidifier les échanges entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, tout en sécurisant les réseaux du quotidien. Il renforcera les liens avec l'agglomération grenobloise et soutiendra l'activité économique et le maintien de l'emploi dans un des territoires français les moins peuplés, largement tourné vers le tourisme, qui souffre d'un enclavement géographique et de difficultés en termes de mobilité.

par rapport aux travaux à mener sur cet axe 21 et son avis sur l'europrojet soutenu- notamment -par les compagnies consulaires des départements concernés.

L'amélioration de cet axe a bien vocation à s'inscrire dans les contrats de plan État-région. Des travaux de mise à 2x2 voies de l'entrée sud de Villeneuve-sur-Lot, la poursuite des études de mise à 2x2 voies de la section La Croix-Blanche-Montbalen,

les logiques de désenclavement, la finalisation d'un certain nombre d'itinéraires ... Je voudrais y apporter ma contribution en évoquant l'A 77.

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a permis l'accélération de la mise en oeuvre du projet de transport, par la création d'un établissement public spécifique chargé de son portage, son financement et sa réalisation. Sa création a été justifiée par l'importance du « projet urbain, social et économique d'intérêt national » visant à « promouvoir le développement économique durable, solidaire et créateur d'emplois de la région capitale afin de renforcer l'attractivité de la région face à la concurrence des autres métropoles mondiales ». Ces objectifs sont équivalents aux priorités identifiées par le Conseil d'orientation des infrastructures, pour « doter la France d'infrastructures performantes au service de l'économie française », en répondant « aux objectifs de transition écologique, de soutenabilité économique et de solidarité » pour la programmation des grandes infrastructures à venir.

Cet amendement vise en conséquence à fixer comme priorité nationale la possibilité de mise en oeuvre de sociétés de financement pour accélérer la réalisation de grandes infrastructures. Leur création a pour but de matérialiser l'engagement commun commun de l'État et de ses établissements publics, ainsi que des collectivités territoriales intéressées par de tels projets, pour assurer, à l'échéance la plus rapide, la réalisation de ces infrastructures, conformément aux préconisations du Conseil d'orientation des infrastructures À ce titre, au regard de l'intérêt structurant du Grand projet du Sud-Ouest pour accompagner le développement démographique et économique du sud-ouest de la France, cet amendement tend l'État crée par priorité un établissement public dénommé Société du Grand projet du Sud-Ouest. Cet outil permettrait en effet d'anticiper le portage financier

? J'ai eu l'occasion de le dire, et cela figure dans l'exposé des motifs, nous travaillons avec les collectivités, s'agissant du GPSO, mais aussi de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, pour examiner dans quelle mesure des ressources locales permettraient, dans le cadre d'une société de projet, d'accélérer la réalisation d'un projet. La contrainte posée, c'est que cette société ne nécessite pas plus de financements que ceux qui sont prévus à l'heure actuelle dans la programmation des infrastructures. Par ailleurs,

Dans une société de projet, on pourrait associer différents projets dans une enveloppe unique. C'est ce que j'ai proposé dans le cas de l'A 31 ce corridor nord-sud très simple, allant de Luxembourg à Nancy,

actualité brûlante, aussi bien sociale que climatique, les manifestations de nos jeunes les vendredis, l'Affaire du siècle, qui a ressemblé plus de deux millions de signataires : tout cela nous appelle à nos responsabilités. Nous avons signé les accords de Paris, et nous en sommes fiers. Il est donc temps d'agir et de mettre en cohérence nos politiques et nos engagements internationaux. Ce n'est pas facile, cela bouscule nos habitudes : c'est justement ce que nous devons faire, car nous sommes attendus. On attend en effet des politiques une véritable révolution. La politique de lutte contre le changement climatique doit devenir une priorité, car les rejets de gaz à effet de serre continuent à augmenter, de 2 % en 2018.

de façon symbolique, ces engagements. Le présent amendement vise ainsi à mettre en cohérence la politique fiscale de la France avec ses objectifs climatiques et à dégager des pistes possibles de nouvelles recettes pour financer le report modal,

et environnemental de mesures fiscales. Il conviendrait aussi d'étudier et de proposer des solutions d'accompagnement pour soutenir les secteurs en difficulté et les aider à réaliser leur transition écologique. Par cet amendement, nous proposons de dresser un état des lieux de l'ensemble des exonérations fiscales dont bénéficie le secteur des transports, tous modes confondus, et de dessiner les perspectives d'une suppression progressive des exonérations fiscales contrevenant aux objectifs climatiques de la France. Nous devons regarder la réalité en face,

Il nous importe de mettre en cohérence la politique fiscale de la France avec ses objectifs climatiques et de dégager des pistes possibles de nouvelles recettes pour financer le report modal,

Il conviendra aussi d'étudier et de proposer des solutions d'accompagnement, pour soutenir de façon vertueuse les secteurs en difficulté, afin de les aider à réaliser leur transition écologique. La suppression des exonérations sur les carburants pourrait par exemple s'accompagner d'une aide

Ce rapport devra comprendre le phasage des travaux et leur financement précisément définis, dans la perspective de la mise en service de ce tunnel prévue en 2030. Il s'agit bien sûr, madame la ministre, d'un amendement de repli. Mes collègues des Alpes du Nord, ceux du Lyonnais et moi-même souhaitons que l'itinéraire du Bas-Dauphiné soit retenu.

Je me sens un peu seule, dans cet hémicycle, pour défendre le département de l'Ain ; je constate que chacun, ici, défend son territoire- c'est bien normal. Mais vous comprendrez

En l'occurrence, l'amendement que je présente avec quelques-uns de mes collègues vise tout simplement à supprimer l'Afitf, l'Agence de financement des infrastructures de transport de

les associations de protection de l'environnement ne participent pas au conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, et c'est probablement un manque. Je prendrai le contre-pied de mon collègue Canevet : l'Afitf est le lieu de création du consensus

pour rendre acceptable un certain nombre d'infrastructures -, alors il faut que les associations y siègent, en amont ; à défaut, on se retrouve, en aval, avec des oppositions et des discussions. La parole est à Mme

qui vient d'être défendu par mon collègue Dantec, vise à ouvrir la gouvernance de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France aux associations de protection de l'environnement. Depuis 2009 et la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, la politique des transports est censée contribuer au développement durable et au respect des engagements nationaux et internationaux de la France en matière d'émission de gaz à effet de serre et d'autres polluants, tout en limitant la consommation des espaces agricoles et naturels. Nous nous devons d'être volontaristes pour protéger l'environnement et conserver la biodiversité. Les politiques de transport sont liées aux enjeux de la protection de l'environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique. En 2018, les émissions de dioxyde de carbone, de CO2, donc, ont augmenté de 2 nous sommes très loin des objectifs fixés par l'accord de Paris. Si l'Afitf coordonne le financement des grands projets d'infrastructures de transport sous la tutelle du ministère de l'écologie, il nous semble pertinent, dans une logique d'urgence climatique, de conformer nos actions aux préconisations des associations de protection de l'environnement,

Il s'agit également, en amont, au niveau de la prise de décision, d'anticiper d'éventuels conflits ou contentieux, dans une logique de démocratie participative et par cohérence avec les objectifs auxquels nous avons souscrit. Aussi ces associations doivent-elles être reconnues comme des membres de droit des instances de gouvernance des autorités ayant pour mission la mise en oeuvre des politiques de transport de notre pays. Quel

Gouvernement pour mettre en oeuvre les projets qui auront été décidés dans le cadre du COI, avec une programmation à respecter et des financements afférents.

par des prélèvements spécifiques au transport routier et qui souhaitent s'assurer que c'est bien au profit du financement de nos infrastructures de transport que ces prélèvements sont effectués.

tant elle nous semble juste pour financer les besoins en investissements en faveur de la mobilité. Nous proposons de créer une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine. Seraient ainsi exonérées de cette taxe les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France. Ainsi, nous tenons compte des spécificités de notre région, puisque, chacun le sait, Paris et les Hauts-de-Seine concentrent une très grande part de l'immobilier de bureaux, totalisant plus de 55 % de l'offre en mètres carrés de bureaux en Île-de-France. La tendance ne fait que s'accentuer, comme le confirment les chiffres de l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise en Île-de-France, avec des emplois qui ne se sont jamais autant polarisés que dans l'Ouest parisien et les Hauts-de-Seine. Cette hyperconcentration participe au déséquilibre en matière de développement économique et territorial, avec une répartition des emplois à l'ouest et de l'habitat à l'est. Cet aménagement du territoire induit de nombreux déplacements et une saturation du réseau existant.

du pays. Quel est l'avis de la commission ? La taxe sur les bureaux, notamment en Île-de-France, est une taxe annuelle qui concerne les locaux à usage de bureaux- locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement. Elle vient d'être réévaluée pour financer le Grand Paris Express. Je ne suis pas favorable à l'empilement de dispositifs additionnels. Plutôt que de créer une taxe nouvelle, essayons de flécher les recettes existantes. La commission émet donc un avis

Cette taxe mettrait à contribution les sociétés et son produit serait affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, l'Afitf. L'institution de cette taxe nous paraît nécessaire au regard de la faiblesse des fonds attribués à l'Afitf. Le rapport annexé au présent projet de loi prévoit en effet une enveloppe de 14,3 milliards d'euros sur cinq ans. Il prévoit également que le budget 2019 de l'Afitf augmente de 10 % par rapport à l'année 2018. Cela peut sembler une avancée de taille, mais, dans les faits, le montant réel des investissements de l'État prévu pour 2019 est inférieur de 200 millions à celui que comporte ce projet De plus, les enjeux contenus dans ce texte sont considérables, puisqu'il s'agit d'apporter des solutions aux territoires qui manquent de ou ont besoin de développer des moyens de transport répondant à l'urgence climatique et environnementale, de renforcer les financements en faveur des transports quotidiens et de développer de nouvelles offres de transport. Ces objectifs sont louables et méritent des financements à leur hauteur. Cette nouvelle taxe permettrait de mener une politique ambitieuse en matière de transport, en répondant aux objectifs précédemment énoncés et en finançant de nouveaux projets. On peut citer l'investissement massif envers les lignes Intercités de nuit, proposé par le groupe CRCE dans un précédent amendement. Par ailleurs, une plus grande mise à contribution des entreprises se justifie pleinement. bénéficieront, en effet, de l'amélioration des services de transport sur le territoire, qui permet de faciliter les déplacements des travailleurs et participe au développement de l'activité économique. Quel est l'avis de la commission ?

amendement vise à instituer une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières. Toutefois, son affectataire n'étant pas précisé, son produit irait par parallélisme au budget global de l'État et au Fonds de solidarité pour le développement et

qui se serait appliquée aux poids lourds sur le réseau routier non concédé, dans le cadre des dispositions de la directive Eurovignette. Dans ses considérants, cette directive indique : « Dans le secteur des transports routiers, les péages, calculés comme des redevances d'utilisation des infrastructures fondées sur la distance, constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durable, puisqu'ils sont directement liés à l'utilisation de l'infrastructure. a déjà été mis en place dans plusieurs pays européens tels que l'Allemagne, l'Autriche ou, plus récemment, la Belgique. Le montant de la redevance aurait été progressif, ce qui aurait permis non une partie des désavantages compétitifs subis par les transporteurs français, mais aussi de favoriser le report modal. Enfin, l'introduction de cette redevance aurait permis, sans préjudice pour les finances publiques, de rétablir une plus grande équité fiscale entre les entreprises de transport françaises françaises et étrangères, en supprimant une taxe à l'essieu discriminante et en permettant à ces mêmes entreprises nationales de dégrever une plus grande part de la TICPE qu'elles acquittent sur leur facture de carburant.

de transport de France, ce qui augmente la capacité de dépense d'un opérateur, le présent amendement aggrave une charge publique au sens de l'article 40 de la Constitution ». Mes chers collègues,

En conclusion, la suppression de la taxe à l'essieu ! l'adaptation des montants de TICPE acquittés par les entreprises françaises ! C'est pourquoi nous proposons de sous-amender l'amendement n° 127 du groupe CRCE, qui vise à faire contribuer davantage les véhicules effectuant des trajets de plusieurs kilomètres, sans pénaliser nos transporteurs nationaux et en réduisant l'empreinte carbone.

ce sous-amendement pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative, dans la mesure où le législateur doit fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature et ne peut renvoyer à un décret la fixation du taux sans l'encadrer autrement qu'en fixant un principe de progressivité en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

c'est que les transporteurs français, encore tout à leur victoire sur l'écotaxe, continuent de dire non à toute nouvelle taxation, y compris à ce mécanisme qui nous semblait séduisant intellectuellement

Deux questions se posent s'agissant des poids lourds. Les coûts des poids lourds français qui font leur plein en France sont

Je voudrais que nous soyons tous conscients de la portée des amendements dont nous sommes en train de débattre. Il s'agit ici d'augmenter la taxe d'aménagement du territoire, qui n'est perçue que sur les autoroutes,

Il est fort dommageable que ce texte ait renoncé à faire contribuer le transport routier à la rénovation de nos infrastructures la création d'une écotaxe poids lourds. Le minimum serait de supprimer les niches fiscales sur les carburants polluants et émetteurs de gaz à effet de serre. Ces financements supplémentaires viendront compléter le budget fragile de l'Afitf. Si nous voulons enrayer le réchauffement climatique, la transition écologique doit également impliquer un report modal, qu'une refonte de la fiscalité doit encourager. La dérégulation économique permet aujourd'hui à des entreprises internationales de réduire à l'extrême les coûts de leurs circuits de production, pour exploiter la faiblesse des normes sociales et environnementales de certains pays. Cela n'est possible que par le faible coût du transport routier, dont les externalités négatives sont assumées par la collectivité. Si ces calculs, qui consistent à séparer les sites de production, d'assemblage et de distribution dans des pays différents, permettent aux directeurs financiers de ces multinationales de s'y retrouver, ils se font en dépit du bon sens et de l'impératif climatique. En plus d'être inadapté aux enjeux écologiques actuels, le transport de marchandises par les poids lourds sollicite les routes et nécessite d'importants et réguliers investissements qui font défaut pourtant à d'autres modes de transports plus vertueux. Le report modal vers des transports moins polluants et la relocalisation vers des circuits courts ne se feront pas sans la taxation du transport routier international traversant la France. Commençons donc par supprimer cette exonération !

de nouvelle taxe. Nous pensons pourtant que celle-ci serait exemplaire et utile, nous permettant d'être plus ambitieux dans nos projets de financements en privilégiant, par exemple, le scénario 3 préconisé par le Cette mesure permettrait ainsi de faire supporter par les véhicules routiers de marchandises la prise en compte d'externalités de ce transport. Le présent amendement vise donc à appliquer en France les dispositions prévues dans la directive européenne Eurovignette III et à orienter les recettes liées à cette redevance vers les transports alternatifs aux transports Il n'y a en effet aucune raison que la France applique avec zèle les directives d'ouverture à la concurrence et qu'elle traîne des pieds sur les directives plus vertueuses écologiquement. Il est important de signaler que cette taxe additionnelle ne handicapera pas le pavillon routier français, puisqu'elle sera exigible à tous les transporteurs empruntant le réseau routier français concerné. Cette internalisation permettra, en appliquant le principe de pollueur-payeur, de réduire les distorsions de concurrence dont bénéficient aujourd'hui les transports les plus polluants, dont la route. Je rappelle les coûts très importants suscités par les externalités de ce mode de transports, la pollution de l'air coûtant à elle seule 101 milliards d'euros et causant 48 000 décès prématurés par an en France. À titre indicatif, les produits de cette redevance seraient de l'ordre de 130 millions d'euros. Ce montant est très loin des impacts financiers des externalités des transports, mais l'introduction de ce principe aurait pour avantage de commencer à permettre la prise en compte des externalités dans les redevances d'utilisation des infrastructures de transport et de doter l'Afitf de nouvelles recettes.

ce transfert de compétences des routes non concédées et des autoroutes a pour unique objectif de permettre à la collectivité européenne d'Alsace d'instaurer un dispositif de régulation du transit poids lourds.

Mon ami et collègue Olivier Jacquin a parlé de celui qui a rédigé cet amendement ; ceux qui l'ont cosigné

et qui a en quelque sorte pris le relais de la commission Mobilité 21, animée et présidée par M. Duron. Pour mener à bien les objectifs inscrits dans ce projet de loi, il est en effet indispensable de disposer de nouveaux outils de pilotage des politiques publiques,

que vous ayez rejeté, madame la ministre, monsieur le rapporteur, toutes nos propositions qui visaient à trouver de nouveaux financements. Pour nous, il convient d'agir sur tous les fronts pour faire du report modal la pierre angulaire des politiques d'investissement dans les transports. Le Conseil d'orientation des infrastructures est l'instance de gouvernance décisive pour assurer le suivi de la programmation des investissements. Il doit permettre de suivre les engagements pris par les pouvoirs publics. Nous regrettons simplement que sa gouvernance ne soit pas précisée. C'est pourquoi nous serons particulièrement attentives et attentifs au décret qui fixera la composition de cette instance. Nous estimons qu'elle doit être ouverte à de nouvelles actrices et de nouveaux acteurs représentant des citoyennes et des citoyens et de l'intérêt général veillant à la lutte contre le changement climatique et à la protection de la biodiversité. Il s'agit des associations, bien sûr, mais également des organisations syndicales qui, par leur engagement au sein du service public, disposent d'une expertise précieuse en la matière. Avec ces précisions, nous soutiendrons cet article.

d'un actif public, d'un bien commun, accumulé quelquefois depuis des décennies, voire plus. Tout le monde connaît l'état de dégradation de certaines petites lignes ferroviaires.

instituer un suivi des investissements réalisés chaque année par cette agence et de la localisation des équipements financés, afin de permettre au législateur d'apporter sa contribution aux orientations de la politique d'investissement de l'État dans les grandes infrastructures de transport. de suivre avec diligence les fonds de l'Afitf et de contrôler leur utilisation.